est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

-pour mesurer les conséquences financières des règles d'approvisionnement de la restauration collective, tant pour les gestionnaires des établissements que pour les usagers. Ce rapport aurait trois objectifs principaux : analyser les surcoûts potentiels ; évaluer le reste à charge pour les usagers et pour leurs familles

? Madame la rapporteur, vous proposez que le Gouvernement remette un rapport au plus tard en janvier 2019. Nous avons déjà prévu une concertation avec les parties prenantes pour la rédaction du décret sur les conditions de mise en oeuvre, telles qu'elles sont prévues dans l'amendement gouvernemental. Cette concertation sera organisée dans le cadre du nouvel organisme qui sera créé d'ici à la fin de l'été, c'est-à-dire le Conseil national de la restauration collective. Je suis très attaché au suivi de l'application de la loi. Nous ferons donc des points d'étape réguliers au Conseil précité. Il y a un enjeu financier, qui est, certes, important, mais il n'est pas le seul. Il faut aussi travailler sur la formation des acheteurs publics, avec l'actualisation de la boîte à outils Localim, que le ministère de l'agriculture a créée, ainsi que sur le développement des projets alimentaires territoriaux, avec l'information sur le maillage territorial de la production et de la distribution. Les dispositions de votre amendement posent aussi une difficulté pratique en fixant l'échéance de ce rapport au 1 janvier 2019. À ce stade, on ne disposera pas du recul nécessaire pour évaluer correctement et objectivement les surcoûts, de même que les problèmes de mise en oeuvre de l'article 11. Pour ces raisons,

La consommation globale de protéines animales est en constante augmentation. L'agriculture mondiale ne pourra pas satisfaire l'ensemble des besoins des populations à la hauteur de l'actuelle consommation des pays développés sans provoquer de nombreux problèmes environnementaux, climatiques et de santé publique.

Le CNRS constate, dans une étude récente, la disparition d'un tiers des oiseaux en quinze ans. En cause, la fin des jachères imposées par la PAC, l'agriculture intensive en monoculture et la généralisation des néonicotinoïdes, qui ont participé amplement à l'effondrement des populations d'insectes- 80 % des insectes ont 35 % du blé européen sont destinés à l'alimentation animale. Plus largement, les animaux sont les premiers consommateurs de céréales en France. Ainsi, en termes de surfaces, l'alimentation animale mobilise en France 14 millions d'hectares de cultures fourragères et 4 millions d'hectares de céréales, oléagineux, protéagineux,

devons rendre la transition des élevages français et l'amélioration du bien-être animal économiquement viables, tout en faisant disparaître les pratiques qui font du tort tant sur le plan environnemental qu'économique. Il est donc nécessaire de diminuer sensiblement notre consommation de protéines animales par habitant. Il ne s'agit pas de ne plus en consommer, mais d'en consommer moins et mieux. C'est pourquoi cet amendement vise, sur l'initiative de France Nature Environnement, à inclure un objectif de rééquilibrage des protéines animales et végétales dans les objectifs de la politique nationale de l'alimentation. l'avis de la commission ? L'article L. 1 du code rural est sans doute l'un des articles fixant des objectifs de politique publique parmi les plus longs et les plus détaillés ; le présent projet de loi l'allonge encore. Il prévoit « d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante ».

du Gouvernement ? Il revient au programme national nutrition santé et au programme national pour l'alimentation, sur la base des données scientifiques, d'adapter et de faire connaître les repères nutritionnels pour promouvoir des choix alimentaires qui soient favorables à la santé et respectueux de l'environnement. Le Gouvernement

Pris à table, à heures régulières, et composés de produits variés, ces repas représentent le socle du modèle alimentaire français. Ce rythme alimentaire est d'ailleurs l'un des facteurs qui permettent à la France de limiter l'accroissement de l'obésité dans la population. Cependant, cet équilibre est menacé, confronté qu'il est à l'importation de comportements alimentaires qui se standardisent à travers le monde. Le petit-déjeuner, par exemple, constitue la base de l'équilibre nutritionnel en France. Il représente en moyenne 20 % de l'apport énergétique total quotidien et il fournit de nombreux nutriments essentiels pour que les enfants en pleine croissance bénéficient de leurs entières capacités physiques et mentales. Pourtant, les chiffres de 2016 du CREDOC sont inquiétants : un enfant sur cinq saute le petit-déjeuner au moins au moins une fois par semaine. Cela entraîne pour toute la journée un décalage dans la prise des repas, ce qui encourage la consommation de et affaiblit les capacités d'apprentissage de l'enfant. Cet amendement vise donc à souligner le rôle central du rythme alimentaire français, pour que ce facteur soit pris en compte dans les programmes d'information et de communication relatifs à l'alimentation et à la santé, notamment à destination des enfants et des adolescents.

pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires ». Cette notion d'équilibre intègre, me semble-t-il, cette dimension de rythme alimentaire quotidien.

Sans cette option, les personnes concernées sont contraintes de manger un repas déséquilibré, ce qui est contraire à l'objectif d'accès à une alimentation de qualité pour tous. Le repas à la cantine étant parfois le seul repas équilibré de la journée, comme on l'a déjà dit, il convient que ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson, ce qui est respectable, aient également accès à un repas de qualité. Cette mesure s'appliquerait aux restaurants proposant déjà au moins deux menus.

Je suis convaincu qu'il est possible d'introduire cette option à coût constant, en agissant par exemple sur la réduction du gaspillage alimentaire. Je précise que je ne souhaite absolument pas attaquer l'élevage. Nombre d'éleveurs réalisent un travail remarquable, essentiel à la vie des territoires, à la structuration des paysages, à l'alimentation de qualité. Je suis également tout à fait conscient de l'efficacité des complémentarités entre productions végétale et animale. Cet amendement ne vise pas à promouvoir la généralisation du véganisme, mais il me semble essentiel de respecter les libertés et les choix alimentaires de chacune et de chacun.

67 % des viandes servies en restauration collective des entreprises, des écoles, des hôpitaux et autres établissements publics et privés sont des viandes importées, d'après les données de l'Institut de l'élevage. Nous le savons, les budgets de la restauration collective étant très contraints, nous servons à nos enfants et aux personnes vulnérables présentes dans les hôpitaux, de la viande importée, la moins chère possible, donc de mauvaise, voire de très mauvaise qualité, produite avec des standards environnementaux et sociaux bien moins exigeants que les nôtres. Pis, dans une perspective de baisse des coûts, il arrive régulièrement que la viande donnée soit de la viande reconstituée. Pendant ce temps, nos éleveurs locaux produisent de la viande de qualité, mais ne trouvent souvent pas un prix rémunérateur dans la restauration collective locale. Proposer un repas végétarien par semaine permettrait de limiter les coûts sur ce repas, sans traumatiser les enfants, et de proposer pour les repas restants une viande de meilleure qualité, produite localement. Cette mesure est pratiquée dans de nombreuses villes. Ainsi,

M. Guillaume Gontard. Cet amendement va dans le même sens que celui de Joël Labbé. Nous cherchons à mener une expérimentation consistant en l'obligation de proposer, chaque jour, un repas de substitution végétalien quotidien dans les services de restauration collective qui propose au moins deux entrées et deux plats principaux distincts. En effet, la législation impose de servir de la viande, du poisson et des produits laitiers à une fréquence définie. Il nous paraît indispensable d'assouplir cette norme pour celles et ceux qui en feraient la demande, en introduisant des menus de substitution végétaliens, dès lors que la capacité du restaurant collectif le permet.

et aller vers une consommation de qualité. Avec vingt kilos de poissons consommés par être humain et par an, les ressources halieutiques sont aussi menacées, 31 % des stocks de poissons mondiaux sont surexploités et 11 % des espèces sont menacées de disparition, notamment celles que nous consommons le plus. Le poisson est tellement essentiel à la survie de l'humanité qu'il faut instaurer une pêche durable et responsable, en laissant les espèces se reproduire, donc diminuer notre ponction sur les océans. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de faire évoluer nos modes de consommation, en vue d'amorcer une diminution de la production carnée et d'en finir avec la surpêche. Il est du rôle du législateur d'accompagner les citoyens déjà engagés dans cette démarche. Une telle expérimentation permettrait également de sensibiliser et d'éduquer les autres, en particulier les plus jeunes, à un type d'alimentation qui comprenne moins de viande, mais qui soit plus local et de qualité, dans l'intérêt des éleveurs. Elle invitera nos cuisiniers à renouveler et à enrichir le vaste répertoire de la cuisine française, en inventant de nouvelles recettes à base de protéines végétales.

Alors que les viandes et les poissons représentent aujourd'hui 20 % du gaspillage alimentaire et 50 % du coût de ce dernier, la législation française impose de servir ces denrées, ainsi que les produits laitiers, à une fréquence définie. Nous proposons, à des fins d'évaluation et d'éducation, une expérimentation d'une durée de deux ans, en introduisant l'obligation d'alternatives végétariennes quotidiennes à base de protéines animales ou végétales dans la restauration collective scolaire publique ou privée. La dimension d'évaluation de cette expérimentation a pour but de déterminer l'incidence de la présence d'options végétariennes sur ce gaspillage alimentaire. La dimension éducative consiste, notamment chez les enfants, à introduire d'autres solutions alimentaires, en raison notamment de l'impact de la surconsommation de viande sur la santé. L'un des enjeux ici est, comme pour bon nombre de points discutés dans ce projet de loi, la santé. De plus en plus d'études tendent en effet à montrer que la consommation de viande en trop grande quantité a, a, ou peut avoir, un impact négatif sur la santé. Elle favorise, par exemple, les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques, comme le diabète de type 2, ainsi que certains cancers. L'ANSES, tout comme le Haut Conseil de santé publique, recommande de ne pas consommer plus de 70 grammes de viande par jour. Consommer de la viande rouge une à deux fois par semaine peut suffire pour assurer les besoins en fer de l'organisme. L'autre enjeu fondamental est celui de l'environnement et de la protection de la planète. Le changement climatique et le respect de la biodiversité, mais également l'augmentation de la population mondiale, nous imposent d'ores et déjà d'explorer des solutions alimentaires alternatives.

incluant des alternatives à base de protéines végétales. Ensuite, il convient de privilégier- je pense que nous en serons tous d'accord -le dialogue au sein des communautés éducatives, plutôt que d'agir par la contrainte. Il faut le savoir, aujourd'hui, les établissements peuvent d'ores et déjà prévoir tous les menus qu'ils souhaitent, notamment des repas végétariens ou l'alternance de poissons ou d'autres protéines, sans pour autant qu'il faille modifier la loi. Enfin, comme M. le ministre l'a souligné tout à l'heure, les repas à la cantine sont, bien souvent et pour de nombreux enfants,

un certain nombre de gens et d'associations n'hésitent pas à caillasser des boucheries, voire des poissonneries. De tels actes sont purement répréhensibles et bien évidemment

de poissons qui venaient d'élevages industriels en Asie du Sud-Est, comme le panga ou d'autres types de poissons qui étaient souvent nourris- on l'a su bien après ! -avec des boues d'épuration.

ni législatif ni réglementaire.

Les petites fermes sont essentielles, car elles maintiennent le tissu rural, sont créatrices d'emploi, valorisent les produits régionaux et sont à la base d'une activité sociale et économique intense. Leur donner une définition légale offrira une transparence bienvenue à tous les consommateurs qui souhaitent favoriser ce mode de

que 15 % des fermes françaises étaient hors-jeu, parce qu'elles n'avaient plus une taille suffisante. Pour ma part, j'estime que les petites fermes peuvent et doivent encore jouer un rôle dans nos territoires, notamment dans le cadre de l'alimentation de proximité.

que leur revenu, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ajouté au chiffre d'affaires est inférieur aux plafonds ci-dessus ; « La moyenne triennale du montant maximum d'aides du premier pilier de la politique agricole commune est de 15 000 euros pour une unité de travail annuel, de 20 000 euros pour deux unités

de la montagne à s'en souvenir.

souvent été objecté qu'il y avait déjà assez de signes de qualité, entre l'agriculture biologique, les labels rouges et les appellations d'origine contrôlée. Or aucun des signes de qualité ou labels actuels ne couvre le terrain de la nutrition et de son lien au mode de production agricole. La démarche portée par Bleu-Blanc-Coeur répond pourtant aux aspirations des éleveurs comme à celles des consommateurs pour les produits de l'élevage français ; il s'agit de croiser une préférence alimentaire nationale avec des qualités intrinsèques améliorées et reconnues. En effet, le lien entre le mode de production agricole, la densité nutritionnelle des produits et le développement de certaines maladies n'est plus à prouver. Des études ont été réalisées par l'AFSSA et l'ANSES à ce sujet. sujet. Cette filière incarne un mode de production figé dans un cahier de charges et contrôlé par un organisme tiers accrédité et indépendant ; c'est une obligation de moyens. Ce mode de production produit une qualité nutritionnelle mesurable et mesurée systématiquement ; c'est une obligation de résultat. Elle est en lien avec une amélioration de la nutrition et de la santé humaine, ce qui contribue, à consommation égale, à atteindre

d'agriculture à intérêt nutrition et environnement » ou « démarche agricole de progrès nutritionnel », qui bénéficierait essentiellement à la démarche privée Bleu-Blanc-Coeur. Ces démarches peuvent tout à fait tout à fait entrer dans le processus de certification au titre d'une démarche valorisante existante. Il ne nous semble pas nécessaire de multiplier les démarches valorisantes

Schillinger. Les acides gras trans industriels sont issus d'un procédé permettant d'avoir des graisses plus faciles à utiliser, qui s'oxydent moins et se conservent donc plus longtemps. On les retrouve aussi, sans le savoir, dans de nombreux produits alimentaires transformés, mes chers collègues, tels que votre croissant de ce matin ou votre quiche surgelée de tout à l'heure. Si cette trouvaille industrielle présente de nombreux avantages fonctionnels, elle comporte aussi un désavantage majeur pour la santé de tous. de la santé a calculé que ces acides gras sont responsables de 500 000 décès par an. Ils augmentent sensiblement le risque de cardiopathie, même à faibles doses, et ont des conséquences importantes sur la survenue de cancers, l'apparition du diabète, le développement foetal et bien d'autres choses encore. L'OMS appelle purement et simplement à leur interdiction d'ici à 2023. Nombre de pays ont déjà agi en ce sens : le Danemark, la Lettonie, les États-Unis, ou encore le Canada, pour ne citer qu'eux. Aussi, je propose que la France aille dans le même sens. Nous pouvons facilement faire un premier pas en les limitant, puis en les supprimant, dans la restauration collective publique en deux ans, afin de laisser aux différents acteurs le soin de s'organiser. Peut-être pourrons-nous, dans un second temps, élargir cette proposition pour les supprimer complètement des aliments achetés et vendus en France.

Ce nouveau label permettra au consommateur d'identifier l'origine des produits et de les différencier des produits importés, notamment du point de vue des normes sanitaires, sociales et environnementales. Cela représenterait un soutien pour les agriculteurs de nos territoires ultramarins.

: La parole est à Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à réintroduire l'expérimentation aux termes de laquelle l'État autorise les collectivités qui le souhaitent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

Il s'agirait d'un engagement fort au diapason avec les voeux de nos concitoyens, qui sont de plus en plus nombreux à être soucieux de leur alimentation. Pour que le consommateur soit en mesure d'effectuer un véritable choix, incitons les collectivités désireuses de participer à cette expérimentation à lui indiquer si les produits sont locaux, surgelés, biologiques, ou encore en boîte. La restauration scolaire, en particulier, répond à une double exigence de maintien de la qualité nutritionnelle des repas et d'information des parents et des enfants.

11 prévoit de « favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation ». Allons dans ce sens et passons aux travaux pratiques ! Quoi de plus ludique pour un jeune enfant ! Quoi de plus ludique pour un jeune enfant qu'un logo doté d'un code couleurs pour se familiariser avec les enjeux de sa santé ?

Mes chers collègues, les fabricants et distributeurs du secteur alimentaire qui s'engagent à utiliser ce logo doivent d'ores et déjà transmettre les données à la section nutritionnelle de l'Observatoire de l'alimentation dont la mise en oeuvre est confiée à l'Institut

Avec le label « fait maison », qui figure dans cet article et qui existe déjà pour la restauration traditionnelle, on risque de ne pas reconnaître ce travail, qui exclut la fabrication en cuisine centrale.

on interdirait l'utilisation de ce label à ceux qui se donnent la peine de confectionner eux-mêmes des gâteaux ou des lasagnes, de travailler les recettes,

La mention « fait maison » suppose aujourd'hui que le plat soit élaboré sur place à partir de produits bruts. Le code de la consommation, dans sa partie

de restauration collective d'ici à 2022. Je me réjouis également que les risques de contamination des produits alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants de cuisson, de réchauffe ou de service soient pris en compte, par le biais d'un rapport qui sera rédigé par l'ANSES. Je soutiendrai d'ailleurs l'amendement de mon collègue Xavier Iacovelli visant l'interdiction de ces outils en restauration collective d'ici à 2022.

cumulés ! Trois phénomènes ont dépassé le seuil d'alerte, à savoir la présence totale de pesticides et celle de deux résidus de désherbants, l'atrazine, qui est un herbicide interdit depuis 2003,

En outre, je m'interroge sur l'interférence de ces substances entre elles, que ce soit l'atrazine, le chlorure de vinyle monomère ou d'autres substances que l'on peut retrouver dans l'eau

les collectivités locales à interdire l'utilisation des contenants en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, en particulier les cantines scolaires. Pour ce faire, il prévue permettra d'évaluer l'incidence sanitaire potentielle, notamment en matière d'exposition à certains perturbateurs endocriniens qui sont suspectés de migrer des matières plastiques dans l'alimentation, du recours à des contenants en verre ou en inox. Elle permettra également de mesurer les surcoûts- l'approvisionnement, la logistique, l'organisation -que cette politique de substitution entraînera nécessairement pour les gestionnaires de services de restauration scolaire. Il s'agit non d'imposer, mais d'agir en concertation, en autorisant les expérimentations. Le libre choix des collectivités

l'utilisation de plastique dans la restauration scolaire ou dans les établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans. Outre que la prolifération des plastiques met en danger l'environnement, notamment dans les mers et les océans, et que la réduction de leur production, comme de leur consommation, est nécessaire, de plus en plus d'études mettent en évidence les risques qu'entraîne leur toxicité. Cette dernière est majeure en raison de la présence de perturbateurs endocriniens. Ainsi, le bisphénol A, reconnu comme « substance extrêmement préoccupante », puis comme perturbateur endocrinien par l'Agence européenne des produits chimiques, est d'ores et déjà interdit dans les contenants alimentaires en France. Mais d'autres bisphénols, notamment F et S, dont la structure moléculaire est similaire, sont toujours utilisés, ainsi que les phtalates, sur lesquels l'Institut sécurité nous alerte., un documentaire diffusé sur Arte, alertait également sur cette question, fondant son contenu sur les propos et les études de plusieurs scientifiques.

Ces perturbateurs endocriniens sont également présents dans les plastiques, y compris alimentaires, au contact direct des aliments. Les réchauffer dans le contenant augmente par ailleurs le risque. Certes, un rapport est prévu pour évaluer les dangers de ces contenants en plastique. Cependant, quelle que soit l'opinion de chacune et de chacun, il est de notre devoir ne pas attendre ses conclusions pour agir. Suffisamment de scientifiques nous alertent pour que nous prenions les devants, ne serait-ce qu'en vertu du principe de précaution. C'est là le minimum que nous pouvons et devons faire : cette mesure relève de la santé publique, et tout particulièrement de celle de nos enfants. L'amendement

Il vise à interdire l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, contenant des substances reconnues comme étant des « perturbateurs endocriniens », au profit de l'utilisation de matériaux inertes et durables au plus tard le 1 janvier 2022.

Certains services de l'État ont d'ores et déjà introduit ce principe de précaution. À titre d'exemple, l'Agence régionale de santé de la région Nouvelle-Aquitaine, dans son guide du mois de janvier 2017, recommande de « privilégier pour la cuisson, la remise en température et le service, la vaisselle en verre, en inox ou porcelaine qui sont des matériaux simples, non identifiés comme sujet aux migrations moléculaires ». Plusieurs collectivités locales se sont également engagées en faveur de la suppression de l'utilisation de barquettes en plastique dans le cadre des services de restauration scolaire.

L'action de l'association Cantine sans plastique France n'y est pas pour rien. Je tiens à saluer son engagement exemplaire dans ce combat sanitaire et environnemental. Elle a d'ailleurs été rejointe par de nombreuses associations de parents d'élèves. Au-delà de l'enjeu sanitaire que présente ce principe de précaution pour les jeunes générations, celui-ci s'inscrit dans la politique de réduction des déchets engagée depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, notamment dans la lignée des interdictions précédemment adoptées dans le cadre de la loi du 17 août 2015,

qu'il n'y a aucun risque à boire de l'eau minérale ou de l'eau de source conditionnée dans une bouteille en plastique. Les bouteilles d'eau en plastique sont composées exclusivement de un matériau chimiquement inerte qui ne migre pas dans l'eau et qui a été validé et approuvé par toutes les agences de sécurité sanitaire des aliments. Contrairement à ce qui a été dit encore récemment, les bouteilles en PET ne contiennent ni bisphénol A, ni bisphénol A, ni dioxines, ni perturbateurs endocriniens. L'eau en bouteille est donc l'un des produits les plus sûrs de notre alimentation, fournie par de nombreux services de restauration collective, notamment pour les publics fragiles, dans les crèches, les hôpitaux ou les EHPAD, les Nous devons laisser le choix à ces établissements de distribuer de l'eau du robinet ou en bouteille. L'eau, qu'elle provienne du robinet ou de sources minérales, joue bien sûr un rôle essentiel pour l'hydratation du corps humain. évidemment essentielle dans le cadre d'une politique de prévention renforcée de lutte contre l'obésité. Mes chers collègues, je vous demande de ne pas pénaliser de façon discriminatoire l'eau minérale naturelle,

que les eaux minérales sont présentes partout sur notre territoire et qu'elles constituent une partie du patrimoine de la France. Monsieur le ministre,

Lutter contre la pollution et garantir la santé alimentaire de nos concitoyens sont des objectifs légitimes, que je partage. Je tiens toutefois à m'assurer que cette mesure n'est pas juste un effet d'annonce et qu'elle repose bien sur une analyse objective et réfléchie. J'aborderai rapidement trois aspects de la question. La pollution due aux plastiques est un fléau mondial qui ne souffre aucune contestation. Toutefois, les bouteilles d'eau minérale en PET sont entièrement recyclables. Reste que les niveaux de tri et de recyclage sont insuffisants. En matière de santé alimentaire, aucune étude réalisée dans notre pays n'a mis en évidence le risque de pollution de l'eau minérale par des perturbateurs endocriniens. On invoque des analyses contraires, réalisées notamment aux États-Unis. Où est la vérité ? Sur quelle étude se fonder ? S'il y a un réel danger, pourquoi ne pas interdire tout simplement, et en toutes circonstances, les bouteilles en plastique ? Qu'en est-il enfin des conséquences industrielles, économiques et sociales de cette interdiction, qui implique de repenser tout le processus industriel d'embouteillage ? Aucune étude d'impact n'a été réalisée. Si nous interdisions les bouteilles en plastique, il faudrait bien les remplacer par un autre contenant.

ce serait le cas dans le département du Nord, où les producteurs devraient se tourner vers la Belgique pour l'embouteillage. Quelles sont les conséquences économiques et sociales, en termes d'emplois, de la disparition des bouteilles en plastique ? Comment relancer une industrie et une production adéquate et suffisante de bouteilles en verres ? ? Toutes ces questions méritent un minimum de réflexion, ce qui n'a pas été fait à l'heure actuelle. La problématique des bouteilles en plastique doit être traitée dans sa globalité, à partir de constats et d'études avérés,

Cet amendement vise également à supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article 11 du projet de loi, qui prévoit de mettre fin à l'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective au plus tard le 1 janvier 2022. Nombre des arguments à l'origine d'une telle mesure se révèlent assez incohérents. point de vue sanitaire, il faut rappeler que l'eau en bouteille, comme cela a été dit, n'a jamais contenu et ne contient pas de perturbateurs endocriniens. Dès lors, introduire une interdiction uniforme sur tout le territoire conduirait à pénaliser les territoires, qui veulent avoir la liberté d'opter

inutile pour la santé, dans un pays où l'eau potable est presque accessible à tous. Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de l'État de New York en mars dernier, et abondamment relayée par la presse française, a mis en évidence la présence de microparticules de plastique dans 93 93 % des bouteilles d'eau examinées, produites par deux cent cinquante grandes marques à travers le monde, dont des marques françaises. Il y en aurait ainsi deux fois plus que dans l'eau du robinet. Il y a un lien, et cette étude le montre, avec certains types de cancer, la diminution de la quantité de spermatozoïdes ou encore l'augmentation de certaines maladies, comme le trouble du déficit de l'attention ou l'autisme. L'influence des microparticules de plastique sur certaines maladies est corroborée par de nombreuses études.

assiettes. Un autre enjeu doit donc nous inciter à limiter le plastique : l'enjeu environnemental. La pollution au plastique est un fléau mondial, et la France n'est pas en reste.

Pour moins polluer, il faut évidemment mieux gérer les déchets, mais en produire moins facilite la réalisation de cet objectif. Rétablissons les porteurs d'eau ! Dans le secteur du recyclage du plastique, la France ne brille pas

ou le service, car le plastique contient des substances reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens. Selon une étude de l'ANSES en 2015, la migration des substances nocives pour la santé du contenant

à rétablir ce que le Gouvernement appelle une « expérimentation au titre de l'article 72 de la Constitution ». Il s'agit d'autoriser les collectivités territoriales qui le demanderaient à interdire les barquettes en plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Je formulerai plusieurs remarques à ce sujet. Premièrement, il faut cesser de prétendre que l'on agit lorsque l'on n'agit pas.

En outre, l'objet de l'amendement me surprend. Le Gouvernement y indique que cette expérimentation permettra d'évaluer l'incidence sanitaire potentielle de ces barquettes. Qu'est-ce que cela signifie ?

et à la remplacer par une interdiction à compter du 1 janvier 2022 des contenants alimentaires en plastique, uniquement lorsqu'ils sont destinés à être en contact avec des aliments chauds ou devant être chauffés et exclusivement dans les cantines des écoles et des établissements accueillants des enfants de moins de six ans. Tant pis pour les autres

vise à interdire l'utilisation des barquettes en plastique dans les cantines pour réchauffer les plats préparés en cuisine centrale. Je n'y reviens pas. Je rappelle que nous avons préféré remplacer l'expérimentation inutile que l'Assemblée nationale avait adoptée par une évaluation complète de l'ANSES. Il s'agit d'évaluer s'il existe des risques de migration de perturbateurs endocriniens vers les aliments. J'ajoute qu'une telle interdiction nécessiterait des investissements importants, notamment une réorganisation des cuisines de ces services. Enfin, nous devons être sûrs de ne pas remplacer ces contenants par d'autres qui seraient nocifs, voire pis

rectifié -, qui visent à supprimer l'interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique dans les services de restauration collective. Ce sujet a été longuement débattu en commission. Nous avons finalement adopté une position que, à titre personnel, C'est pourquoi je souhaite en dire un mot, si vous me le permettez, madame la présidente. J'entends les arguments économiques avancés par ceux qui relaient les préoccupations légitimes de l'industrie des eaux minérales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais proposé en commission de repousser la date de cette interdiction à 2022, au lieu de 2020.

faut savoir que, quoi que nous fassions, nous irons inévitablement vers un modèle plus sobre en ce qui concerne la consommation de nos ressources. Il va falloir arrêter de produire autant de plastique en France. Je rappelle que notre pays produit plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques par an et que seuls 20 % de ces déchets sont aujourd'hui recyclés. Nous pouvons supprimer cette interdiction aujourd'hui, mais, je vous préviens, demain, c'est la Commission européenne qui la décidera. Eh oui ! Tel est d'ailleurs le sens de la proposition de directive sur les déchets marins qu'elle a présentée à la Je pose la question : avons-nous vraiment besoin de bouteilles d'eau en plastique dans les cantines ? Il existe tout de même des solutions de remplacement, comme les carafes en verre ou en inox, que nous avons tous connues lorsque nous étions au collège. La vérité, c'est que nous savons que nous n'en avons pas besoin.

que, depuis 2016, le tri à la source et la collecte séparée sont obligatoires pour les entreprises produisant plus de 1 100 litres de déchets par semaine et pour les administrations publiques et les établissements publics. Ce tri concerne aussi le papier, les métaux, le plastique, le verre et le bois. La quasi-totalité des services de restauration collective a donc l'obligation de procéder à ce tri, ce qui limite considérablement la portée de ces deux amendements. La commission émet donc un avis défavorable

dans une abondante littérature scientifique, notamment par l'ANSES et par le Conseil général de l'environnement. Une agence régionale de santé a même évoqué le principe de précaution dans son rapport.

d'or. Aberration écologique, économique et sociale, 420 millions d'euros d'argent public vont être mobilisés

visent à supprimer l'interdiction de l'utilisation des bouteilles en plastique dans la restauration collective à partir de 2022. Comme l'a expliqué le rapporteur pour avis, ces amendements ont reçu

Les dispositions de cet amendement pourraient paraître anecdotiques. Pourtant, il n'y a pas de petite pollution par les plastiques : nous devons donc nous montrer intraitables en matière de risques sanitaires et environnementaux provoqués par les matières plastiques.

est la plus touchée par cette pollution. En mer du Nord, 95 % des fulmars trouvés morts avaient du plastique dans leur estomac. Un peu partout, nombre d'espèces ingèrent les micro-fragments plastiques, en les confondant avec le phytoplancton ou le zooplancton, et en crèvent. Des études montrent que deux cent soixante espèces animales ingèrent ces fragments et sont étouffées par eux. De fait, le problème des plastiques, c'est qu'ils ne se dégradent pas, mais se fragmentent en morceaux infiniment petits. Selon l'expédition MED, on dénombre dans certaines zones de la Méditerranée autant de micro-fragments plastiques que de plancton par mètre carré ! Plus généralement, il arrive que l'on dénombre jusqu'à 900 000 micro-déchets plastiques par kilomètre carré dans certains secteurs,

pour la croissance verte, a interdit l'utilisation des sacs plastiques à usage unique. Seront interdits en 2020 les gobelets et assiettes en plastique, sauf ceux qui sont compostables. L'Union européenne propose d'interdire une dizaine de produits plastiques, dont ceux que je viens de citer. Il est vrai qu'elle est la dix-huitième pourvoyeuse mondiale de détritus plastiques. Il me semble donc souhaitable que la France, qui a déjà pris un peu avance dans sa législation, complète la liste des produits déjà interdits, en y ajoutant les pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons. En fait, il s'agit de cibler les dix premières sources de déchets marins, qui sont des objets plastiques

plus la densité des microparticules plastiques dans l'environnement augmente, plus la probabilité est grande qu'elles finissent par s'accumuler dans les chaînes alimentaires et, pourquoi pas, jusque dans nos assiettes et nos estomacs. Cela ressemblerait à un retour à l'envoyeur. Très bien

pour les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation de saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Quel est l'avis de la

par un trop grand nombre de demandes. Je m'attendais bien à ce que le Gouvernement invoque la séparation des pouvoirs pour proposer la suppression de ces dispositions. Certes, l'ANSES est un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, mais en aucun cas la disposition visée ne remettra en cause l'autorité de l'exécutif sur cette agence. Il s'agit simplement de permettre aux commissions permanentes du Parlement de saisir l'ANSES en vue de la réalisation d'une étude, afin que nous puissions être éclairés lorsque nous élaborons la loi. À titre d'exemple, une telle disposition permettrait à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de demander une étude sur les effets de l'invasion des sargasses aux Antilles,

d'abord, le Gouvernement fait planer le risque d'une censure constitutionnelle. J'invite chacun à demeurer humble et à se garder de présager de la position des juges de la rue de Montpensier, surtout dans un domaine Le Conseil constitutionnel s'est pour l'heure borné à interdire qu'un organe parlementaire chargé de l'évaluation des politiques publiques puisse, sur le seul fondement du règlement de l'assemblée, bénéficier du concours d'experts placés sous la responsabilité du Gouvernement. Nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. De plus, il n'est pas question de modifier la gouvernance de l'ANSES ou de la placer sous la cotutelle du Gouvernement et du Parlement. Le Parlement n'aura pas autorité sur l'ANSES ; il disposera simplement d'un moyen de conforter son expertise et son information. Ensuite, il y va de l'expertise du Parlement et de sa capacité d'évaluation. Nos collègues de l'Assemblée nationale ne cessent de réclamer davantage d'expertise. Pourquoi ne pas recourir à celle qui existe déjà et dont la compétence comme l'indépendance sont reconnues par tous ? En En proposant la suppression de l'article, le Gouvernement semble vouloir réduire la capacité d'information du Parlement. En l'état actuel du droit, presque tout le monde peut saisir l'ANSES, sauf le Parlement répondra peut-être que les associations de défense des consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au conseil d'administration du Fonds ainsi que certains réseaux sanitaires, ont un intérêt à agir. Mais qu'en est-il du Parlement, chargé de faire la loi ? Enfin, le Parlement a déjà confié à l'ANSES la réalisation de certains travaux. Ainsi, l'article 125 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages confie à l'agence la réalisation d'un bilan sur les bénéfices et les risques liés aux usages des néonicotinoïdes. Plus largement, combien de lois contiennent des articles demandant des rapports au Gouvernement ? J'émets donc un avis défavorable

: La parole est à Mme Angèle Préville. Sur la proposition de Mme la rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté, à juste titre, un amendement visant à permettre aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation de saisir l'ANSES.

les commissions permanentes sont amenées à examiner des textes législatifs, l'OPECST est un organe qui n'a pas à connaître de projets de loi ; c'est un organe de contrôle qui assure l'interface entre le monde scientifique et le monde politique et un organe d'information du Parlement. En tant que tel, il a la possibilité d'auditionner l'ANSES, par exemple. Réservons la possibilité de saisir l'agence aux commissions, qui seront amenées à trancher pour telle ou telle option dans le cadre de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi. J'émets donc un avis défavorable.

M. Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous proposons de rétablir cet article supprimé par la commission des affaires économiques du Sénat, en y apportant des modifications, afin d'améliorer la transparence de l'information aux usagers. Nous avons élargi le dispositif en ajoutant les établissements accueillant des enfants de moins de six ans. Sans phase d'expérimentation, nous rendons obligatoire l'affichage des menus mentionnant l'origine des produits, ainsi que le nom des producteurs. Il s'agit ici de répondre à une attente sociétale forte, tout en promouvant les producteurs locaux et les producteurs responsables ; nous revenons ainsi au débat que nous avons eu précédemment sur l'information des consommateurs dans la restauration collective. Les

par Mme la rapporteur, qui prévoyait que les services gestionnaires des services de restauration scolaire, universitaire et des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans soient tenus d'informer et de consulter régulièrement les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

selon l'origine des aliments et des produits, de leur composition nutritionnelle, ainsi que des mesures prises pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Actuellement, l'article L. 230-5 du code rural précise que ces établissements sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Cet amendement vise donc à accompagner cet objectif en fixant des points d'étape, afin de mesurer l'avancée des progrès réalisés par les établissements, ainsi que les efforts encore à mener pour améliorer la qualité des repas servis. Il nous semble s'intégrer totalement dans la logique de ce texte, à savoir améliorer la qualité de l'offre alimentaire et engager les acteurs dans une démarche de progrès, de transparence et de suivi.

Cet amendement vise à supprimer le contrôle de constitutionnalité par le Gouvernement de l'extension de l'article 11 à la restauration collective privée. Il n'appartient pas au Gouvernement de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives adoptées par le Parlement.

à M. Roland Courteau. Les menus sans viande se développent de façon croissante dans la société française. Cette pratique saine pour la santé et l'environnement est appelée à progresser, dans la mesure où une consommation carnée moins importante est indispensable. Cet article, intégré par voie d'amendement en commission, limite le développement de ces menus, en interdisant aux produits sans viande de faire référence à un steak ou une saucisse, des termes normalement associés à des produits d'origine animale. Autrement dit, un steak végétal ne pourra plus se vendre sous le nom de « steak », alors que l'emballage indique clairement qu'il ne contient pas de viande. Le consommateur, lorsqu'il achète ce produit, le fait en toute connaissance de cause, et pour la bonne raison qu'il ne contient pas de viande. Il n'est donc Il n'est donc en aucune manière trompé. Ces produits jouent également un rôle important dans la transition d'un régime carné à un régime sans viande. Interdire les dénominations communes de « steak » ou de « saucisse » est un non-sens environnemental et sociétal. Cet amendement a pour objet de permettre aux consommateurs de consommer moins de viande, avec des produits permettant une transition efficace vers un régime végétarien.

La séance est suspendue.